qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'une part, et qu'une candidature pour siéger au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'autre part,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

En premier lieu, cet amendement vous invite à tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe de 3 % sur les dividendes, censure qui a pour effet de dégrader le solde budgétaire de 4,1 milliards d'euros en 2018. En effet, la décision du juge constitutionnel conduit à majorer les remboursements et dégrèvements prévus au titre de l'exercice 2018 de 4,7 milliards d'euros, soit la différence entre les 5 milliards de décaissements prévus et les 300 millions initialement provisionnés dans le PLF. Les contributions exceptionnelles et additionnelles créées dans le cadre de la première loi de finances rectificative viennent, quant à elles, accroître de 600 millions d'euros les recettes d'impôt sur les sociétés en 2018. En second lieu, les amendements adoptés par le Sénat conduisent à améliorer le solde budgétaire de 785 millions d'euros.

et à la minoration des droits de partage pour un coût total d'environ 2 milliards d'euros. À cela s'ajoutent diverses mesures de minoration des recettes fiscales ou tendant à réduire ou à supprimer des plafonds de taxes affectées.

Le vote de cette mesure vise explicitement à participer de l'équilibre de la réforme du logement prévue dans le PLF. Le Gouvernement accepte cette proposition de compromis du Sénat et vous propose d'en tirer les conséquences par anticipation sur le vote de la seconde partie, en augmentant les dépenses du budget général de 700 millions d'euros. En effet, pour que cette hausse de TVA puisse se faire au bénéfice des organismes de logement social, comme le souhaitent les auteurs de cet amendement, il serait nécessaire, en seconde partie, d'augmenter de 700 millions d'euros les crédits consacrés aux aides à l'accès au logement portées par la mission « Cohésion des territoires », ce que le Gouvernement proposera ultérieurement dans le cours

Concernant plus précisément ce dont nous sommes responsables, c'est-à-dire l'incidence des mesures que nous avons adoptées en première partie, les votes du Sénat permettent d'améliorer le solde de l'État de 785 millions d'euros.

où elle s'inscrit dans une stratégie où le taux du livret A a été maintenu. Il y a donc un peu de marge de manoeuvre, ce qui rend cette mesure possible. Si nous avons fait ce choix, c'est d'abord et avant tout parce que nous souhaitons que le Sénat dise que l'article 52,

je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. Je rappelle au Sénat que, conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1août 2001 et à l'article 47, alinéa 2, de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté ». J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat, décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de cinq minutes pour ces explications de vote, à raison d'un orateur par groupe, l'orateur des sénateurs non inscrits disposant de trois minutes.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi de finances est la deuxième étape du moment clé que nous vivons ; moment clé où, pour les cinq années à venir, le Gouvernement installe le cadre de sa politique.

La deuxième étape, c'est la partie « recettes » de ce projet de loi de finances. Les choix qui en découlent ne répondent pas à la grande tâche qui devrait être celle de démocratiser la République, c'est-à-dire la réponse à l'intérêt général. Si votre politique, monsieur le secrétaire d'État, ne répond pas aux attentes des Françaises et des Français, c'est d'abord parce qu'ils ne l'ont pas décidée. La France est prise en otage en otage par le traité européen de 2012, celui de la « concurrence libre et non faussée », traité d'ailleurs non ratifié par le peuple et qui verrouille la souveraineté budgétaire de notre pays. Détaillons les faits. de l'impôt sur le revenu, vous procédez à un relèvement du barème estimé à 1,1 milliard d'euros. Cela n'entraîne aucune augmentation de pouvoir d'achat pour 98 % des Français, mais 440 millions d'euros en plus pour les 2 % des ménages les plus riches. Quant au prélèvement forfaitaire unique, il représente 1,4 milliard d'euros de gains, toujours pour les mêmes 2 %. Et pour les Français modestes ? Vous leur imposez- nous venons d'en parler -une hausse de la TVA dans les HLM 140 euros par an et par locataire. Et à la demande des banques et des marchés financiers, vous fiscalisez l'épargne logement ! Concernant la taxe d'habitation, vous prenez les Français en étau : d'un côté, la droite sénatoriale maintient un impôt injuste

d'étonnant à ce que vous ayez refusé nos propositions d'augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Nous en avons débattu ici : les collectivités territoriales sont une nouvelle fois des variables d'ajustement pour servir l'appétit de la finance. Parlons enfin de l'impôt de sur la fortune. Là, c'est le récit du hold-up des marchés financiers et des banques qui se dévoile ouvertement. Version majorité présidentielle : la réforme coûte 4,2 milliards d'euros aux contribuables. Version majorité sénatoriale : la réforme

Ce projet, dicté par l'Europe de la finance, c'est celui de la classe des milliardaires, qui s'enrichit toujours plus. Oui, elle s'enrichit ! Arrêtez de parler de l'exil fiscal et des malheurs des riches ! Personne ici n'a pu nous contredire

Une nouvelle fois, on assiste à un désengagement des plus fortunés de l'effort de solidarité nationale et de financement des services publics de la nation. Supprimer l'ISF, quelle belle idée nouvelle !

C'est au nom de ce principe que vous avez refusé notre proposition d'un impôt sur le revenu plus progressif, plus juste pour les classes moyennes et populaires. C'est aussi au nom de cette idée de l'argent que vous avez refusé de mettre à contribution le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et le crédit d'impôt recherche, lesquels, conjointement, représentent 27 milliards d'euros de pertes de recettes pour l'État, grâce à l'omerta de Bercy. Monsieur le secrétaire d'État, vous ne mettez pas la République en marche, mais l'égalité à l'arrêt. Vous refusez le projet d'une France en commun ; c'est pourquoi nous voterons contre cette loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, parmi les causes de la défiance de nos compatriotes à l'égard de la chose publique et du monde politique, il en est une, bien connue c'est le manquement à la parole donnée. Les Français attendent qu'on leur dise la vérité et qu'un cap soit fixé. Le projet de loi de finances répond secrétaire d'État, ce budget et la trajectoire dans laquelle il s'inscrit traduisent votre volonté de respecter nos engagements européens. Il réduit la dépense publique et le déficit, respectivement de 0,7 point et de 0,3 point de PIB. Nous souscrivons à cette ligne politique. Pour que la voix de la France soit entendue, pour que la France soit crédible, elle doit d'abord respecter ses engagements européens. Les Allemands, pour les respecter, la sécurité, à la lutte contre le terrorisme, à la délicate question des migrants, à la transition écologique, à l'emploi dans une économie mondialisée, où le dumping social l'emporte souvent sur le respect des êtres humains -, nous ne pouvons pas les relever seuls face au monde. C'est avec nos partenaires européens que nous réussirons. C'est pourquoi nous devons donner un nouvel élan à la construction d'une Europe forte, qui allie réalisme économique, humanisme et justice sociale. En second lieu, ce budget traduit des choix courageux, l'objectif étant de réussir simultanément le pari du désendettement et celui de la relance de l'emploi par l'activité économique. Notre économie doit être au rendez-vous de la révolution numérique et de la transition énergétique : il y va de la capacité de notre pays à créer les emplois de demain. ce point de vue, votre objectif d'orienter le capital et l'épargne vers le financement de nos entreprises et la création d'emplois. Bien sûr, il s'agit d'un pari sur l'avenir, pour tenter de gagner la bataille de l'emploi. Mais tant d'autres solutions ont depuis si longtemps montré leurs limites. Toutefois, nous considérons que le dispositif que vous proposez consistant à supprimer l'ISF pour créer l'IFI ne répond pas à cet objectif. D'un côté, des capitaux ne seront plus taxés alors qu'ils ne seront pas investis dans l'économie réelle. De l'autre, l'immobilier locatif sera taxé, alors que les investissements qui y sont liés soutiennent notamment le secteur du bâtiment et la création d'emplois dans tous les territoires de France. les collectivités et la fiscalité locales, malgré tout ce qui a pu être dit, dans l'ensemble, votre budget préserve la capacité des collectivités à poursuivre leurs missions en 2018. Et le pacte de contractualisation que vous leur proposez va dans le bon sens Mais, vous le savez, les élus ont besoin de visibilité, et il faut garantir des ressources sur la durée à tous les niveaux de collectivités, comme vous le faites, d'ailleurs, pour les régions, auxquelles sera désormais attribuée La suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages dès 2018, à laquelle je reste personnellement favorable, a suscité l'inquiétude des élus locaux, non sur le principe consistant à alléger les charges qui pèsent sur les familles modestes, mais quant à la pérennité des ressources des collectivités. L'engagement, pris par le Président de la République devant les maires de France, d'une remise à plat de la fiscalité locale, avec la probable suppression pour tous de la taxe d'habitation à

avec plus de conviction encore qu'il ne le faisait au début de l'examen du texte. Certes, on peut noter quelques avancées, mais elles sont bien peu nombreuses. Ainsi, nous pouvons nous réjouir de l'exclusion de certaines compensations d'exonération du périmètre des variables d'ajustement.

S'agissant toujours des opérateurs de l'État, et plus particulièrement des chambres de métiers et de l'artisanat, le maintien du déplafonnement des contributions des chefs d'entreprise permet de maintenir les fonds en faveur de la formation des artisans, comme le prévoit la loi Travail de 2016. Dans un domaine bien différent, nous nous réjouissons que le régime fiscal applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne soit simplifié par application d'un seuil unique d'exonération d'impôt à 3 000 euros. nous sommes parvenus dans le cadre d'un groupe de travail de la commission des finances, constitue une mesure de clarification nécessaire. Enfin, un amendement visant à doter les collectivités chargées de l'élaboration des schémas environnementaux, notamment des plans climat, nous paraît aller dans le bon sens ; il en va de même pour le maintien du dispositif ZRR

Du point de vue des collectivités locales, le dégrèvement proposé pour 2018 nous convient. Mais il faut comprendre notre position comme un engagement à se lancer sans tarder dans une réforme en profondeur de la fiscalité locale.

lourde de sens, s'appliquant à un texte déjà par trop favorable aux plus favorisés de nos concitoyens. Je rappelle d'ailleurs que cette baisse de 3 milliards d'euros suit d'autres baisses, de 3 milliards d'euros en 2016 et de 2 milliards d'euros différentes baisses ayant été décidées par le précédent gouvernement. Nous regrettons également vivement le vote d'un amendement créant une nouvelle tranche d'imposition sur le revenu à 5,5 %. Cela fera entrer de nouvelles personnes, les plus pauvres, dans l'impôt. Faut-il rappeler que tous participent déjà à l'effort public, par d'autres types de prélèvements que l'impôt sur le revenu, notamment la TVA et la CSG ? À l'issue de l'examen de cette première partie, le projet de loi de finances est plus que jamais celui de l'injustice fiscale. Il était déjà très favorable aux contribuables les plus aisés, et la majorité sénatoriale n'a fait que renforcer ce travers. Elle a ainsi choisi, sous couvert de redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes, de relever l'avantage fiscal lié au plafonnement du quotient familial. Ce faisant, elle s'adresse en réalité aux ménages appartenant au décile le plus élevé des revenus. Et puis, elle a finalement réalisé un vieux rêve : elle a enfin trouvé le courage de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune sans d'ailleurs ne gager aucunement cette perte de ressources. Pour notre part, nous ne partageons en rien la confiance du Gouvernement quant à l'effet positif à attendre de la limitation de l'ISF à l'immobilier ou de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Ces mesures, profondément inégalitaires, ne constituent que des allégements massifs de fiscalité. Nul ne peut garantir qu'ils permettront d'assurer un quelconque dynamisme à l'économie française. Le Gouvernement ne nous a apporté aucun élément concret en ce sens durant les débats. Plus que tout, ces mesures sont choquantes, au vu des efforts qui sont demandés en parallèle au monde du logement social, aux collectivités territoriales. Elles sont choquantes aussi quand on diminue, pour des raisons plus idéologiques que réellement étayées, les budgets de politique de l'emploi. Je le disais en introduction, au-delà d'une mesure sur le pouvoir d'achat des Français que nous pouvons, avec quelques réserves, partager, nous ne saurions approuver le triptyque suppression de l'ISF, prélèvement forfaitaire unique, impôt sur la fortune immobilière et, bien entendu, encore moins le volet « recettes » du projet de loi de finances tel qu'il a été voté par la majorité sénatoriale.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les débats autour de la première partie du projet de loi de finances touchent à leur fin. Je tiens à saluer l'endurance du rapporteur général et du président de du président de la commission des finances, uniques, ainsi que celle des ministres, nombreux, qui ont joué leur rôle avec une patience, une rigueur et une pédagogie qui honorent, je le crois, notre assemblée. Nos débats ont d'abord permis l'adoption de mesures catégorielles bienvenues, notamment en faveur des biocarburants les plus respectueux de l'environnement, des PME et des agriculteurs. La fiscalité est un outil qui, utilisé avec modération et responsabilité, permet d'encourager les secteurs en difficulté et de soutenir les filières d'avenir. Notre assemblée, guidée par la vigilance du rapporteur général, en a fait bon usage. Nos débats ont également permis de clarifier les positions de chacun et d'exprimer de véritables choix politiques. Les trois grandes réformes du projet de loi de finances ont ainsi été abordées avec vigueur, et chacun a pu exprimer sa position. Certains ont jugé que le Gouvernement allait trop loin ; d'autres qu'il fallait l'aider à franchir un pas supplémentaire ; d'autres, enfin, qu'il fallait donner du temps au temps. Le résultat en est que nous examinons aujourd'hui un texte dont la lettre, mais également l'esprit ont été profondément modifiés. La réforme de la taxe d'habitation, mesure de pouvoir d'achat emblématique de ce projet de loi de finances, est annulée. Le prélèvement forfaitaire unique est conforté et amélioré. L'ISF est totalement supprimé. S'il existait un équilibre dans ce budget, il a été rompu. Le « budget pour les riches » que certains annonçaient risque d'être devenu ici même une réalité. Entendons-nous bien : nous sommes favorables à la suppression de l'ISF, qui est un impôt antiéconomique. Je tenais à le préciser pour ne pas faire peur à nos collègues du groupe communiste. Nous sommes favorables à une refonte globale de la fiscalité locale, qui ne doit cependant pas demeurer un serpent de mer prétexte à l'inaction. Enfin, nous sommes favorables au prélèvement forfaitaire unique, qui simplifie la fiscalité et nous rapproche du niveau de prélèvement européen. Néanmoins, le jusqu'au-boutisme d'un côté et l'attentisme de l'autre ont produit un texte déséquilibré, qui fait plus de gagnants chez les millionnaires et plus de perdants chez les classes moyennes. Surtout, en écartant la nuance, ce texte passe à côté de l'occasion d'améliorer qualitativement les différentes mesures proposées. Tout d'abord, conduite dans les conditions politiques et institutionnelles actuelles, la suppression pure et simple de l'ISF nous fait manquer l'occasion d'aménager et de sécuriser l'impôt sur la fortune immobilière. Alors que ce gouvernement a enfin le courage de supprimer les trois quarts de l'ISF, le Sénat fait primer l'affichage d'un volontarisme décalé sur l'opportunité d'accompagner et d'affiner, en responsabilité, une mesure qui va, quoi qu'on en dise, dans le bon sens.

Ensuite, sur la taxe d'habitation, nous sommes tous d'accord ici sur le fait qu'une réforme globale de la fiscalité est nécessaire. Nous arrivons au bout d'un modèle qui est essoufflé et qui doit être remplacé. Le Président de la République et le Premier ministre s'y sont engagés, bien que les modalités de la future concertation demeurent floues. Nous avons tort, néanmoins, de prendre pour prétexte à l'inaction le grand soir fiscal qu'on nous annonce les premières victimes seront, comme souvent, les classes moyennes, qui trouveront dans le présent budget bien peu de lots de consolation ou de raisons d'espérer pour l'avenir. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Indépendants - République et Territoires, dans sa grande majorité, s'abstiendra sur le texte qui nous est proposé.

Comme chaque année, ce marathon fiscal est riche en débats techniques et politiques, et nombre de mesures ont été examinées. La Chambre haute représente une étape particulière du parcours législatif, puisque la majorité diffère de celle de l'Assemblée nationale et que, du fait de ses spécificités, elle porte davantage son attention sur ce qui concerne directement les terroirs et les territoires. Particulièrement attentif à ces sujets, le groupe du RDSE a, comme chaque année, apporté sa pierre à l'édifice. Je me félicite de l'adoption d'un certain nombre d'amendements, tels que- d'amendements, tels que- dans la lignée du radical Joseph Caillaux -le rétablissement de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui doit rester un impôt citoyen, mais aussi le référencement de biocarburants, des amendements sur les ressources des départements, des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce ou encore sur le Fonds de prévention des risques naturels et majeurs. Ce projet de loi de finances est un baptême du feu pour le nouveau gouvernement, en particulier pour vous, monsieur le secrétaire d'État. Comme on pouvait s'y attendre, les débats se sont concentrés sur des réformes emblématiques, comme le dégrèvement de la taxe d'habitation. Sur ce sujet complexe, la majorité sénatoriale a décidé de rejeter la réforme proposée. S'il est vrai que celle-ci ne réglera pas tous les problèmes ni toutes les injustices, on ne peut, pour autant, pas maintenir la fiscalité locale en l'état, car les bases restent profondément obsolètes et injustes. En revanche, je tiens à saluer l'adoption des amendements concernant l'imposition des services de plateformes en ligne de type Amazon ou Airbnb, car ces activités, par une évaporation des bases taxables, constituent une concurrence déloyale pour les acteurs plus traditionnels des secteurs du commerce et du tourisme. L'amendement sur la territorialisation de la contribution climat-énergie répond, comme le souhaitaient les auteurs d'autres amendements- je pense notamment à mon collègue Ronan Dantec -, à des attentes fortes des collectivités, en particulier les régions et les intercommunalités, qui sont, dans les territoires, les acteurs incontournables de la transition écologique. L'article 12, sur la réforme de l'ISF, a également suscité beaucoup de débats. L'imposition du patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier, constitue un point focal de notre débat économique. Toutefois, les montants en jeu, s'ils ne sont pas négligeables, ne représentent qu'une petite partie des ressources. Pour les recettes de l'État et l'équilibre des finances publiques, les sujets liés à la TVA, à l'impôt sur le revenu ou encore à la fiscalité énergétique semblent beaucoup plus déterminants. Je regrette que le débat sur la taxation allégée des produits de première nécessité, protection des personnes âgées et couches pour les nourrissons, débat souhaité par mon collègue Jean-Marc Gabouty, n'ait pas rencontré autant d'attention qu'il le méritait. Nous tâcherons de revenir sur ces questions, qui restent préoccupantes pour les personnes et les établissements concernés. Enfin, je souhaite aborder les ressources des collectivités. Comme d'autres de mes collègues, je salue la suppression de la CRFP, la contribution au redressement des finances publiques, appliquée sans discontinuer sous le précédent quinquennat. Toutefois, des inquiétudes demeurent sur le sort qui sera réservé aux collectivités, notamment la réforme de la fiscalité locale, mais aussi la contractualisation prévue dans la loi de programmation, pour laquelle la commission mixte paritaire n'a pas encore été réunie. Nous avons, lors de l'examen de cette première partie,

même si les collectivités sorties du classement cette année continueront de bénéficier de certains avantages jusqu'en 2020. Nous estimons que le classement actuel en ZRR ne cible pas suffisamment les territoires les plus ruraux et qu'il devrait s'établir à l'échelle du département, et non des intercommunalités. Enfin, nous avons défendu le développement économique des territoires, notamment l'artisanat, par le biais du soutien aux réseaux des chambres de métiers. Et, clin d'oeil aux fêtes de fin d'année, nous avons également soutenu la trufficulture ! Très bien ! Après ces explications, et comme mon groupe soutient globalement la politique de ce gouvernement, mais tient à garder sa liberté de vues et de vote, nous ne pouvons pas souscrire à toutes les modifications adoptées par la majorité sénatoriale, malgré quelques avancées.

dans quelques minutes, le Sénat se prononcera sur la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Nous voici donc arrivés au milieu du gué. Notre vote ne sera pas une surprise : nous adopterons la première partie telle que modifiée par la majorité sénatoriale, mais aussi par l'ensemble du Sénat, tant les votes ont dépassé les clivages sur un grand nombre de sujets. Depuis que j'ai l'honneur de siéger parmi vous, j'ai appris que c'était là la marque de fabrique du Sénat : l'intérêt général et le travail de fond priment les postures. Notre groupe a donc adopté les mesures qui lui semblaient aller dans le bon sens, tout en les complétant parfois. Ainsi, nous avons inséré des clauses anti-abus dans le nouveau système d'imposition forfaitaire des revenus mobiliers, afin d'éviter de possibles transferts massifs, dans un souci d'optimisation fiscale, des revenus du travail vers les revenus du capital. Nous avons également réécrit l'article réformant l'impôt de solidarité sur la fortune en supprimant l'impôt sur la fortune immobilière, après avoir démontré le caractère productif d'un grand nombre d'investissements immobiliers et l'importance économique du secteur privé du logement. Le gouvernement auquel vous ne reconnaissait d'ailleurs aucune vertu à cet impôt dans l'étude préalable annexée au projet de loi en le qualifiant d'impôt de rendement, maintenu à des fins budgétaires. Le Sénat a également souhaité rééquilibrer la répartition de l'effort fiscal. Notre assemblée a ainsi rétabli la tranche de l'impôt sur le revenu à 5,5 %, supprimée en 2014, reporté la réforme de la taxe d'habitation, dont le caractère injuste du fait des valeurs locatives non harmonisées aurait reposé, de manière encore plus injuste, sur seulement 20 % des contribuables, et relevé le plafond du quotient familial à 1 750 euros par demi-part. Nous avons également ajusté la trajectoire carbone pour adapter l'ambition écologique, que nous partageons, aux réalités économiques. La TICPE ne doit pas être une « vache à lait ». Nous rejetons une fiscalité écologique punitive. Nous pensons que les recettes de cet impôt doivent être utilisées au plus près des citoyens, notamment en donnant aux collectivités les moyens de mettre en oeuvre leur plan climat-énergie. Nous avons restauré une franchise d'impôt de 3 000 euros pour tous les Français qui perçoivent des revenus complémentaires grâce à l'économie des plateformes collaboratives. Ainsi, nous entendons libérer encore davantage l'initiative entrepreneuriale individuelle. Notre économie doit en effet s'adapter aux évolutions et aux défis de la révolution numérique. Pour y parvenir, nous avons souhaité encourager l'innovation des PME. Le Sénat, sur des initiatives venant de toutes les travées, a ainsi voté un amortissement accéléré pour les robots, logiciels et imprimantes 3D, ainsi qu'un suramortissement de 40 % des investissements des PME. C'est dans cet esprit d'accompagnement de la transformation numérique de notre économie que nous avons adopté à l'unanimité un dispositif de solidarité financière des plateformes numériques en cas de signalement de fraude à la TVA liée à leurs activités de commerce en ligne.

que c'était un facteur de complexité et d'illisibilité. C'est la preuve que la refonte de notre fiscalité locale est devenue un impératif. Monsieur le secrétaire d'État, le Sénat entend jouer pleinement son rôle et vous accompagner au plus vite dans cette réforme structurelle, dans un esprit de responsabilité. Animé d'une volonté de compromis transpartisan, le Sénat a travaillé à trouver une solution sur la question des bailleurs sociaux. Une première avancée a été trouvée cet après-midi ; nous resterons cependant vigilants. C'est dans ce même esprit de responsabilité que nous aborderons la seconde partie du projet de loi de finances. À la suite des votes du Sénat, le solde public est amélioré de 785 millions d'euros, mais nous souhaitons aller encore plus loin. La majorité sénatoriale présentera ainsi un certain nombre de mesures d'économies. En effet, nous pensons que l'effort de réduction de la dépense publique doit être engagé dès à présent, afin de profiter du contexte économique plus favorable, et non pas reporté en fin de quinquennat. Monsieur le secrétaire d'État, le Sénat est au rendez-vous de ce début de quinquennat : il exprime des convictions et est une force de propositions. Il est utile au débat, et nous espérons que le Gouvernement, mais aussi l'Assemblée nationale sauront reconnaître l'essentiel du travail que nous aurons accompli à l'issue de la seconde partie, que nous aborderons dès demain en séance publique. En attendant, le groupe Les Républicains votera la première partie du projet de loi de finances tel qu'il a été enrichi.

remercie, monsieur le président. Si l'équilibre est visuellement amélioré, c'est au prix de renoncements que le groupe La République En Marche ne cautionne pas. Notre groupe s'abstiendra : rejeter la première c'est couper court à la discussion ; l'adopter, c'est accepter les bouleversements du texte. La suite est d'ores et déjà connue : nous ne voterons pas l'ensemble du projet Nous avons assisté à des manoeuvres de report visant à toujours tout retarder alors que la France ne peut plus attendre les transformations. Très bien ! Combien de temps encore faudrait-il abuser de la patience des Français ? Combien de temps encore faudrait-il retarder l'application du projet du Président de la République ? Je déplore avant tout la suppression pure et simple de l'article prévoyant l'exonération pour 80 % des foyers de leur taxe d'habitation. Il est étrange de dire que l'on souhaite soutenir les familles en favorisant les plus aisées avec le quotient familial et de refuser d'alléger leur charge fiscale le lendemain. En fait, ce que nous propose la majorité sénatoriale, c'est reculer, mais ne jamais sauter ! Le Président de la République, dans son discours de clôture devant le congrès des maires, a pourtant indiqué que cet engagement était le premier pas d'une refonte plus globale de la fiscalité locale. Le groupe La République En Marche sera pleinement mobilisé sur ces chantiers, avec l'ensemble des autres groupes, car il n'est pas toujours bon d'ajouter de la division à la complexité. Sur d'autres travées de l'hémicycle, fiscalité du patrimoine, affirmant que ce n'était pas le bon moment. Mais ce que nous voulons, c'est justement renforcer la meilleure santé économique de notre pays dès à présent. Et je passe sur ceux qui voulaient reporter la trajectoire de la tonne carbone ou diluer la fiscalité écologique sous de fallacieux prétextes. Manoeuvres dilatoires, propos contradictoires ... À droite, nous avons vu une longue série d'orateurs venir faire amende honorable, comme en pénitence, s'excusant de n'avoir pas eu le courage de supprimer l'ISF. Mais Comme disait Oscar Wilde : « Il ne faut jamais trop se critiquer soi-même, les autres ont tendance à vous croire. » En l'occurrence, on vous a crus ! Vous avez donc proposé de supprimer totalement l'IFI pour vous faire pardonner, mais sans compenser nettement la

Taxe d'habitation, ISF ... Le projet est plus défiguré que le portrait de Dorian Gray. Le groupe LREM s'oppose totalement à cette version sénatoriale. Mais, voter contre la première partie, ce serait refuser la suite des débats. Or nous les attendons pour voir quelles sont les économies que vous proposez enfin ! Vous n'allez pas être déçus ! Ceux qui nous proposent des baisses de fiscalité supplémentaires sont en général les mêmes que ceux qui refusent les économies en seconde partie. Nous en avons eu un avant-goût

Nous avons également interrogé notre procédure budgétaire : à l'occasion des nombreux amendements sur les carburants, la question de la portée juridique de nos débats a été clairement posée. Nos méthodes de travail doivent évoluer dans le sens d'une plus grande évaluation ; cela a été souligné. Nous avons également amélioré la fiscalité sur l'économie collaborative et l'économie numérique. Nous avons Nous avons encore beaucoup à faire pour simplifier notre système fiscal, qui s'éloigne de l'épure du jardin à la française, comme en attestent les nombreuses dépenses fiscales. C'est dans ce sens qu'il faut travailler, celui d'une évaluation raisonnée, d'un travail méthodique et d'une amélioration de la lisibilité de notre système fiscal. Dans cette voie raisonnable,

Le scrutin est ouvert.

Monsieur le ministre d'État, ministre de l'intérieur, depuis les attentats de 2015 en France, la prévention de la radicalisation est devenue une priorité. Pour assurer la sécurité des Français, le Gouvernement a complété l'arsenal juridique et mis en place un renforcement des moyens et des effectifs dans la police, la justice, l'armée et les services de renseignement. Dans ce cadre, un diplôme universitaire de prévention devait être lancé en janvier dernier à l'Institut de droit et d'économie Paris-II Assas de Melun, en Seine-et-Marne. D'abord reporté en septembre dernier, le décret que devait prendre Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre, n'est toujours pas paru. Les enseignements organisés pour l'obtention de ce diplôme intitulé « Faits religieux, droit et société » visent à donner des clefs de compréhension sur des thèmes tels que la laïcité, le fait religieux en France, le droit des cultes et les institutions. Ils visent plus particulièrement la professionnalisation des aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires de toutes confessions, mais ils sont également ouverts à d'autres publics tels que les DRH d'entreprises, les cadres de la fonction publique hospitalière, les personnels de l'éducation nationale, les élus locaux, tous confrontés au phénomène de radicalisation. D'ores et déjà, cinquante candidatures parmi les centaines reçues ont été retenues, pour vingt-cinq places prévues pour la première session. Monsieur le ministre d'État, il est évident que notre pays ne peut se permettre de se passer d'une initiative qui renforcerait un dispositif destiné à prévenir et détecter la radicalisation sur le territoire. Je vous demande donc de bien vouloir nous exposer votre position sur cette formation, très attendue par le directeur de l'Institut universitaire, mais également par les aumôniers et les candidats déjà inscrits. La

le diplôme auquel vous faites allusion s'inscrit dans le cadre de la politique que nous menons avec Mme Vidal, ministre de l'enseignement supérieur. Il vise à améliorer la formation de tous ceux qui, ministres du culte, aumôniers, agents publics, acteurs locaux, sont confrontés à des problèmes liés au fait religieux, à la laïcité ou à la radicalisation. Cette politique s'est mise en place à partir du décret du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique, qui permet de consolider leur formation. Ce texte Ce texte rend obligatoire, pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés, l'obtention d'un diplôme après le suivi d'une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Un arrêté du 5 mai 2017 prévoit une liste de diplômes agréés. Aujourd'hui, une vingtaine de formations sont disponibles partout sur le territoire, y compris en formation à distance : 350 personnes y sont inscrites cette année, dont un tiers sont des ministres du culte. Le dispositif fonctionne donc bien. Le diplôme « Faits religieux, droit et société » de l'Institut de droit et d'économie de Paris-II Assas ne fait pas, à ce jour, partie de ce dispositif, car il n'a pas été demandé d'agrément. Évidemment, si cette demande avait lieu,

Les demandes d'asile continuent d'augmenter. On dénombre pour 2016 un peu plus de 53 000 personnes déboutées, et la situation ne s'arrange pas en matière d'éloignement des personnes en situation irrégulière. Le Président de la République et le Gouvernement ont affirmé à plusieurs reprises leur ferme volonté de lutter contre l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, le Président de la République est en déplacement en Afrique.

de façon à ce que la demande d'asile soit traitée sur place. Cela afin d'éviter de revivre sur notre territoire, comme sur le territoire européen, des situations telles que celles de Calais, de Paris ou ailleurs.

rapport. Je partage vos sentiments sur l'effort à faire en matière de politique d'immigration. Nous devons à la fois

de 4,5 millions d'euros. Oui, nous nous soucions de l'éloignement. Nous allons créer, d'ici à la fin de l'année, 400 places

de l'agriculture. Les représentants des pays membres de l'Union européenne ont trouvé ce lundi un accord concernant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour cinq ans. Votée à la majorité qualifiée, cette décision n'est pas conforme à ce qu'avait défendu la France. Le Président de la République a fait savoir qu'il a demandé au Gouvernement de prendre « les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France [ ...] au plus tard dans trois ans ». Je pense, monsieur le ministre, que l'ensemble des parlementaires ici présents est favorable à ce que l'on recherche des alternatives au glyphosate. La profession agricole elle-même soutient le lancement d'un contrat de solution pour remédier à cette utilisation. solution pour remédier à cette utilisation. Est-il concevable qu'on fasse subir, pendant deux ans au moins, une nouvelle distorsion de concurrence à nos agriculteurs, alors même, je le rappelle, qu'ils traversent une crise sans précédent, qu'un sur trois gagne moins de 350 euros par mois, et que le Président de la République avait pris l'engagement, durant sa campagne électorale, de stopper toute forme de surtransposition européenne en matière agricole ? Eh oui quelle est la cohérence du Gouvernement quand, dans le même temps, il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui permettra d'importer en France des produits contenant des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays ?

vous posez une question sur un sujet extrêmement sensible. Vous l'avez dit, hier, dix-huit États membres de l'Union européenne ont voté pour le renouvellement pour cinq ans de l'autorisation d'utilisation du glyphosate. La France a voté contre. Le soir même, le Président de la République a précisé le cap pour la France : sortir du glyphosate dès que les alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans les trois ans.

Ce qui est attendu du Gouvernement, c'est qu'il mobilise tous les acteurs, ensemble, vers la sortie du glyphosate : les chercheurs, pour trouver des alternatives- l'INRA y travaille déjà - ; les services de l'État, pour réfléchir à des restrictions d'usage efficaces et rapidement opérationnelles ; les producteurs, sans lesquels rien ne sera possible et dont les contraintes doivent être pleinement prises en compte dans la construction de solutions nouvelles ; les experts sanitaires, car il est indispensable de sortir des divergences entre l'OMS et les agences européennes sur la dangerosité réelle du glyphosate. C'est au vu de tout cela, ainsi que du chemin qui aura été parcouru d'ici à trois ans, que l'on saura s'il y a surtransposition ou non. Prenons deux hypothèses. Si tous les experts convergent pour reconnaître une dangerosité extrême, l'Union européenne sera sans doute sensible aux enjeux de santé publique. Si les utilisateurs réussissent

pour mobiliser la recherche et les instituts techniques, mais aussi pour accompagner nos agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques agronomiques. Vive

L'Union européenne vient d'autoriser pour cinq ans supplémentaires l'utilisation du glyphosate, créé par Monsanto et dont on s'interroge sur les effets cancérogènes probables. Les consommateurs sont inquiets et s'expriment de plus en plus vivement sur la qualité des produits alimentaires et leur impact sur la santé. Les agriculteurs, eux, contestent la décision de la France d'interdire l'utilisation du glyphosate sur son sol dans trois ans au plus tard, comme cela a été annoncé hier par le Président de la République. Malgré de nombreuses études, il est quasi impossible de savoir, à ce jour, si le glyphosate et ses additifs sont toxiques pour l'homme ou pas. Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'OMS, a annoncé des effets cancérogènes probables, alors que l'Agence européenne de sécurité des aliments est arrivée à une conclusion inverse. Différentes études individuelles aboutissent, elles aussi, à des évaluations contradictoires. Au regard de ces diverses conclusions, il semble indispensable de revoir le processus d'évaluation de ces substances. Je vous remercie, madame la ministre, de bien vouloir m'indiquer si les trois ans annoncés seront suffisants pour mener à bien des études fiables et si nous avons la capacité de trouver prochainement des alternatives à l'utilisation de ce produit. En outre, comment la France envisage-t-elle d'agir auprès de la Commission européenne afin d'élaborer une stratégie de sortie rapide de l'utilisation du glyphosate ?

le vote intervenu hier en faveur du renouvellement pour cinq ans de l'autorisation du glyphosate est pour nous une déception. Nous avions voté contre. Notre mobilisation a toutefois été utile, puisque nous partions d'une première demande de la Commission en faveur d'un renouvellement pour dix ans. Vous avez raison de le dire, le fait que les analyses européennes ne classent pas le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme, alors que le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, le fait, pose la question de la confiance de l'évaluation européenne. Aujourd'hui, cette confiance est entamée. Il faut donc agir. C'est pour cela que Nicolas Hulot a demandé Hulot a demandé au Conseil des ministres de l'environnement, dès le 13 octobre, de revoir en profondeur l'évaluation européenne des substances chimiques, afin d'aller vers plus de transparence et d'indépendance. La Commission présentera une communication sur ce sujet ; nous en discuterons avec les États membres et le Parlement européen. Nous restons déterminés. Sur le plan national, le Président de la République a demandé au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France, dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans. Certaines alternatives existent déjà et devront être généralisées. D'autres restent encore à développer. Le Gouvernement est pleinement mobilisé et conscient de la nécessité d'accompagner les agriculteurs dans cette transition. Les ministres de l'agriculture et de l'alimentation et de la transition écologique et solidaire feront prochainement des propositions à cette fin.

Ayant quitté récemment mes fonctions de président d'une agglomération qui a pu bénéficier des crédits TEPCV, je peux attester de l'effet de levier considérable de ce dispositif. Un dispositif d'autant plus déterminant pour mon territoire qu'il est en reconversion post-industrielle minière et confronté à une triple nécessité remédier à des pollutions multiples des sols, reconquérir des friches industrielles et développer des modes alternatifs de production et de consommation des énergies. Je salue l'annonce de l'inscription de crédits supplémentaires, à hauteur de 75 millions d'euros, qu'une loi de finances rectificative devra toutefois confirmer, et je remercie M. le ministre des propos rassurants qu'il a tenus lors de son audition par la commission de l'aménagement du territoire

Je souhaiterais donc connaître les intentions et positions du ministre sur plusieurs points. Tout d'abord, la circulaire du 26 septembre induit un traitement purement administratif et mécanique, qui risque de mettre fin à des projets qui seraient pourtant extrêmement bénéfiques pour les territoires concernés. Le ministre entend-il laisser à certains projets la possibilité d'être financés sur la base d'une évaluation de leur intérêt pour le développement local, et ce au-delà même d'irrégularités de la procédure, et dès lors que les collectivités sont engagées dans le cofinancement des projets ? Ensuite, quelle est la position du ministre sur la proposition de l'association AMORCE, soutenue par ailleurs par la grande majorité des associations de collectivités, d'instituer une dotation territoriale climat pérenne ? Enfin, quel est le calendrier gouvernemental concernant la mise en place des futurs contrats de transition écologique et quel serait le niveau de financement dont pourraient bénéficier les collectivités au titre de ces contrats ? S'agira-t-il de « l'autre cadre de financement » mentionné dans la note du 20 novembre ? Auquel cas, la fixation du calendrier n'en serait que plus urgente. La parole

sur les contrats de transition écologique. Le Premier ministre Édouard Philippe m'a demandé de retenir 15 à 20 territoires démonstrateurs pour l'année 2018. Il s'agira de territoires français très différents : littoraux comme montagnards, ruraux comme urbains, métropolitains comme ultramarins. La liste de ces territoires sera arrêtée arrêtée à horizon du mois de janvier. La doctrine précise de ces contrats sera fixée lors de la Conférence nationale des territoires du mois de décembre. J'ai été auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale

Je me doutais qu'il y aurait une réaction. Bien évidemment, nous ne manquerons pas d'étudier cette proposition dans le cadre de la généralisation des contrats de transition pour l'année 2019. La

consacrées à la prévention et à la lutte contre la prostitution, violence extrême à l'encontre des femmes. Doute et vigilance quand l'essentiel repose sur les associations qui luttent contre ces violences et qui n'ont pas les subventions indispensables. Doute et vigilance quant à la création d'unités hospitalières pour la prise en charge psychotraumatique psychotraumatique des victimes dès l'année prochaine, alors que le budget de la sécurité sociale et celui des hôpitaux sont en berne. Doute et vigilance quand le grand absent de ce plan est le monde du travail : rien pour lutter contre les inégalités salariales, suppression des CHSCT

aussi, sur le glyphosate. Ce seul mot peut soulever des tempêtes. Entre querelles d'experts et surenchère des lobbies, le consommateur n'y voit plus clair. Pourtant, il est précisément au centre de ce débat européen, car il est question de santé publique. Comme il y a un doute, notre responsabilité est d'appliquer le principe de précaution, mais le législateur que nous sommes n'a aucun critère objectif pour appréhender la dangerosité ou non de ce produit. En effet, depuis 2015, l'Organisation mondiale de la santé a émis des avis contraires sur cet herbicide ; pour l'Agence européenne de sécurité des aliments. Comment s'y retrouver ? Car, autour de ce débat scientifique, on retrouve des enjeux économiques et financiers énormes.

qu'il n'y aurait aucune surtransposition des normes. Vous avez expliqué votre position, mais je crains que le délai de trois ans ne soit trop court. Ce délai de trois ans est-il suffisant pour trouver, grâce à la recherche, un produit de substitution ? Des agriculteurs se sont déjà tournés vers des pratiques vertueuses qu'il faut encourager, mais une large majorité n'est pas encore sur cette voie. Car, derrière les effets d'annonce, derrière les postures, il y a la réalité d'une filière et d'une consommation qui passe majoritairement par la grande distribution, et où l'origine des produits est mondiale. Au-delà de l'interdiction, il est donc primordial de mettre en place une véritable politique de traçabilité. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord ? Cela vous semble-t-il possible dans un délai aussi court ? Par exemple, qui assurera qui assurera au consommateur français que le pain qu'il achète n'est pas issu de farine de blé provenant du Canada, où le glyphosate a été reconduit pour quinze ans ?

le savez, a clairement cherché un possible. Elle devait dégager une majorité qualifiée au sein des vingt-huit États membres pour les prochaines années. Cette majorité qualifiée, elle l'a trouvée hier sur la durée du renouvellement de

Républicains. Ma question s'adresse à Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le chef de l'État s'est exprimé samedi 25 novembre, lors d'un discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, déclarée « grande cause du quinquennat », au cours duquel il a annoncé ses « trois priorités » : « l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité », « un meilleur accompagnement des victimes » et « un renforcement de l'arsenal répressif On ne peut que souscrire à ces trois axes prioritaires. L'objectif est vertueux, car, même si les rapports et la situation des hommes et des femmes ont évolué ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire en faveur des femmes, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. On sait que la situation des femmes est parfois difficile, du fait des violences sournoises qu'elles subissent et de la banalisation de ces violences. Dans certains quartiers, les femmes ne peuvent plus sortir seules, ni porter de jupe ou de pantalon, par crainte de recevoir une bordée d'injures. La mise en cause de la parole des femmes victimes de ces agissements et l'impunité des agresseurs sont intolérables. Cette situation n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Madame la secrétaire d'État, évoquant les missions de votre secrétariat d'État, vous avez déclaré ceci : « La politique de l'égalité femmes-hommes doit prendre en compte les spécificités des territoires. En d'autres termes, on n'apprécierait pas de la même façon l'égalité entre les femmes et les hommes selon l'endroit où l'on est. Ma question est simple : existe-t-il des territoires de la République où les droits des femmes ne seraient pas les mêmes et pas les mêmes que ceux des hommes ? La parole Je me suis déjà expliquée sur cette phrase, mais je vous remercie, madame la sénatrice, de me donner l'occasion de le refaire. Quand ai-je dit que les politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes devaient tenir compte de la spécificité de chaque territoire ?

aucunement mention des territoires perdus de la République. Je déplore, et j'ai déploré pendant des mois, l'instrumentalisation odieuse qui a été faite par l'extrême droite de cette phrase sortie de son contexte. Je vous remercie donc, une nouvelle fois, de m'avoir posé cette question, qui me permet de répondre très clairement

Madame la ministre, je souhaiterais vous alerter sur une situation qui préoccupe de nombreux élus de métropoles, notamment ceux du département du Puy-de-Dôme autour de Clermont-Ferrand. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a permis la création de quinze métropoles entre janvier 2015 et juillet 2016. La loi de finances pour 2017 a doté les métropoles créées avant janvier 2017 d'une enveloppe de 150 millions d'euros, qui a servi à financer les quinze pactes métropolitains. Ce statut répondant à un réel besoin en matière d'organisation et de renforcement des territoires, notamment après la réduction du nombre des régions, sept nouvelles métropoles seront créées en janvier prochain, dont celle autour de Clermont-Ferrand. Or le projet de loi de finances pour 2018 ne prévoit aucun fonds destiné au lancement et au bon fonctionnement de ces métropoles, ce qui crée de fait un grand déséquilibre avec celles créées avant 2017. Pour Clermont Auvergne Métropole, c'est un manque à gagner d'environ 10 millions d'euros, soit un coup d'arrêt ou une ambition territoriale revue à la baisse. Que pouvez-vous répondre, madame la ministre, aux élus dont les territoires ont été reconnus plus tardivement comme métropoles et qui ne bénéficieront pas des financements promis ? Ainsi, sept agglomérations- Dijon, Metz, ... Ah ! ... Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Tours et Clermont-Ferrand -se voient offrir un statut de métropole de seconde zone. Dans un gouvernement où l'innovation et l'entrepreneuriat sont valorisés, comment expliquez-vous ce désengagement de l'État sur un sujet qui touche à la fois à la valorisation de l'économie locale, au développement de la recherche et à la promotion internationale de nos territoires ? La parole

Le Président de la République l'a rappelé lors du congrès des maires, il existe des métropoles d'envergure européenne et mondiale et d'autres qui sont non pas de seconde zone, ...

un pacte État-métropoles a été signé avec certaines d'entre elles. Naturellement, les opérations lancées seront financées jusqu'à leur terme. De manière générale, les nouvelles métropoles vont bénéficier d'un statut protecteur équivalent à celui des métropoles existantes. Ce statut est inscrit dans la loi quant aux compétences essentielles qu'elles exercent sur leur territoire. Pour le calcul des dotations de fonctionnement de l'État, notamment la dotation d'intercommunalité, ce statut les protège et leur est favorable, comme il protège les autres métropoles. À partir de 2018, la méthode de calcul sera identique à celle utilisée pour les autres métropoles. concerne les dotations d'investissement, elles seront évidemment éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local, pour contribuer au financement de leurs projets structurants, au même titre que les métropoles déjà créées avant le 1 janvier 2018. Ce financement est donc commun à toutes les métropoles. Enfin, le soutien de l'État s'adaptera aux enjeux de chaque métropole. Nous demanderons aux préfets de soutenir en priorité, notamment, les investissements transformateurs mis en oeuvre dans une logique de réciprocité et de complémentarité entre les territoires, comme il en a déjà existé deux exemples en France, à Toulouse et à Brest. La parole

Hier, les syndicats ont appelé à la grève dans le réseau d'enseignement français à l'étranger pour protester contre la réduction de 33 millions d'euros du budget alloué à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'éducation fait partie des priorités du Président de la République. Le ministère de l'éducation nationale a obtenu une augmentation de son budget de 1,3 milliard d'euros, quand l'AEFE a, quant à elle, vu sa subvention baisser de 33 millions d'euros, soit 10 % de son budget. À la rentrée scolaire, les établissements scolaires conventionnés ont été informés que, au lieu des 6 % de rétrocession habituels sur les écolages, ce chiffre passerait à 9 %, ce qui signifiait que, au 1 janvier 2018, les frais de scolarité seraient mécaniquement augmentés. Le réseau AEFE est l'un des fleurons du rayonnement de l'éducation française à l'étranger, et 60 % d'élèves étrangers le fréquentent. Le Président de la République est intervenu devant les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger le 2 octobre et s'est engagé à ne pas modifier les subventions à l'AEFE en 2018 et 2019. Il s'est fait applaudir sur cette promesse, alors qu'en réalité la baisse venait d'être décidée ... La confirmation de cette baisse pénaliserait les lycées et les familles et entraînerait une perte d'influence pour notre pays et le déconventionnement de nombreux établissements. Quelle est l'intention du Gouvernement ? Souhaitez-vous supprimer l'AEFE et qu'il n'existe plus d'établissements conventionnés dans le réseau ?

est sans équivalent chez nos partenaires à travers le monde. J'en parle volontiers, car tous mes enfants y ont été scolarisés. Ce réseau est au service de nos compatriotes installés à l'étranger. C'est aussi un outil d'influence, puisqu'il assure la diffusion de notre langue, de notre culture et de nos valeurs auprès d'un public constitué, vous l'avez dit, aux deux tiers d'élèves de nationalité étrangère. C'est la première priorité budgétaire de notre diplomatie d'influence, qui lui consacre 60 % de son budget, et cela va le rester. En 2017, il a été demandé à l'AEFE de prendre sa part de l'effort collectif de réduction des dépenses. La subvention pour cette année a été diminuée à hauteur de 33 millions d'euros. Une série de mesures ont été prises. Je souligne que les suppressions de postes ne toucheront pas d'enseignants en cours de contrat, que le plafond d'emplois est préservé, ce qui permet le recrutement d'agents en contrat local, et que les subventions aux établissements pour renforcer leur sécurité sont maintenues. Dans ce contexte, j'entends, comme vous, les inquiétudes qui s'expriment aujourd'hui. Je voudrais rappeler ici l'engagement du Président de la République, qui a salué, devant l'Assemblée des Français de l'étranger, le travail de l'AEFE et de ses personnels et qui a confirmé que ses crédits seraient préservés en 2018 et en 2019. Au-delà, nous devrons écrire ensemble l'avenir du réseau français à l'étranger en travaillant avec l'AEFE,

Madame la ministre, il est évidemment plus facile de couper les budgets des Français de l'étranger, qui ne viendront pas bloquer Paris ... Le réseau est en danger, et il nous paraît indispensable de rétablir le budget initial de l'Agence, afin qu'elle puisse accomplir sa mission. On assiste à une diminution constante des sommes consacrées au rayonnement de la France à l'étranger, alors que notre Président de la République se déplace dans le monde entier en essayant de faire croire le contraire.

dans son discours de samedi dernier. C'est une excellente initiative que de consacrer l'égalité entre les femmes et les hommes « grande cause du quinquennat » ou encore de décider la sanctuarisation des crédits dédiés. Cependant, certains regrettent que l'exécutif tente de faire passer des vessies pour des lanternes, qu'il dissimule certains reculs et qu'il essaie, comme trop souvent, de faire croire que rien n'avait été fait avant l'avènement de La République En Marche. Félicitons-nous, tout d'abord, que vous vous inscriviez dans la continuité du cinquième plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette cause dépasse les clivages et les partis. Il est donc juste de reconnaître le travail effectué par les ministres de droite et de gauche qui vous ont précédée. Venons-en maintenant aux lanternes. Le budget interministériel dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes atteindrait désormais 420 millions d'euros, contre 313 millions l'an dernier. L'augmentation est-elle si importante ? Plusieurs journalistes, militants et parlementaires ont calculé que ce n'était pas le cas. M. Macron a en réalité ajouté au montant de ce budget des actions qui n'étaient pas comptabilisées comme telles l'an dernier : par exemple, 65 millions d'euros au titre des chèques emploi pour la garde d'enfants ou 26 millions consacrés aux places en centres d'hébergement. J'ai aussi évoqué des reculs. Il y a les conséquences concrètes de la baisse des emplois aidés- je pense, par exemple, à l'antenne du planning familial dans mon département de Saône-et-Loire. Il y a aussi la baisse de 300 000 euros des crédits consacrés par la justice et la police

Je n'ai jamais dit que notre action avait commencé avec La République En Marche. J'ai au contraire rappelé, à chaque fois, à quel point le combat et le mouvement féministes s'inscrivaient dans une longue histoire, combien les droits des femmes étaient récents au regard de l'histoire de l'humanité,

produit d'un système. Il faut donc des crédits interministériels et transversaux pour lutter contre le système qui produit ces violences et pour les éradiquer.

En effet, elle n'a entraîné aucune économie budgétaire, ainsi que la Cour des comptes vient de le confirmer dans un récent rapport. En revanche, en raison de leur étendue démesurée, ces régions n'ont plus aucune proximité avec le terrain. Ainsi, la région Grand Est est-elle plus grande que la Belgique tout entière, laquelle est pourtant divisée en trois régions. De même, elle est plus étendue que le total des trois allemands qui sont nos voisins. nos voisins. Pour réduire le fameux millefeuille territorial de manière pertinente, il aurait fallu s'inspirer de la réforme du conseiller territorial lancée par le Président Sarkozy. Celle-ci conservait les anciennes régions, qui étaient à taille humaine. En revanche, les départements avaient vocation à se dissoudre en leur sein, ce qui supprimait une couche du millefeuille précité. Aujourd'hui, un fort mécontentement s'exprime dans plusieurs anciennes régions. C'est notamment le cas en région Alsace, qui, comme vous le savez, a une très forte identité et, de plus, fonctionnait de manière remarquable avant qu'elle ne soit engloutie dans le magma du Grand Est. Les Alsaciens ont raison de réclamer le rétablissement d'une région Alsace qui absorberait les deux départements pour former une collectivité alsacienne unique. Le gouvernement Valls a imposé une décision brutale, sans aucune concertation, lorsqu'il a décidé de fusionner d'office les anciennes régions, qui, pourtant, ne lui demandaient rien.

le principe d'un référendum permettant aux Alsaciens et aussi aux Lorrains de s'exprimer sur l'éventuel rétablissement de leur ancienne région ? La parole

le Président de la République s'est engagé à ne pas faire de « big-bang territorial », c'est-à-dire à ne pas revenir sur les réformes lancées au cours des cinq dernières années.

des forces vives du territoire. Si cette condition est remplie, notre droit permet de faire beaucoup de choses. Des délégations de compétences entre collectivités et des rapprochements de départements pourront être entrepris pour répondre aux souhaits des élus et de la population, mais cela dans le cadre de la région Grand Est.